La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 6 novembre 2024 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n’y a pas d’observation ?… Le procès verbal est adopté. Mes chers collègues, par lettre en date du 6 novembre, M. Guillaume Gontard, président du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, demande l’inscription à l’ordre du jour de l’espace réservé à son groupe, le jeudi 19 décembre, de la proposition de loi en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie. Pour l’examen de ce texte, nous pourrions prévoir une discussion générale de quarante cinq minutes. En outre, nous pourrions fixer le délai limite pour le dépôt des amendements de séance au jeudi 12 décembre à douze heures, et pour les inscriptions des orateurs des groupes au mercredi 18 décembre à quinze heures. Par ailleurs, les jeudis 14 novembre et 19 décembre, nous pourrions débuter l’examen des textes dans le deuxième espace réservé dès la fin du premier, si celui ci se terminait avant

pour la France ? » Dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes question disposera alors à son tour du droit de répartie pendant une minute. Monsieur le ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, une fois que celui ci aura retrouvé une place dans l’hémicycle.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un nouveau cycle institutionnel s’amorce pour l’Union européenne. Le moment est propice pour réfléchir ensemble à la politique européenne qu’il faut engager pour les cinq prochaines années et sur l’influence

Désormais, la donne politique a changé : il faut compter avec deux nouveaux blocs puissants, les droites souverainiste et populiste, qui constituent les troisième et quatrième groupes au Parlement européen, en lieu et place des libéraux de Renew Europe et des Verts sous la précédente législature.

Les politiques industrielles agressives conduites par Pékin et Washington nous mettent parfois dos au mur. La défiance de nos populations envers la construction européenne et le populisme qui s’en nourrit ne peuvent plus rester sans réponse, sauf à se résigner à voir les extrêmes conquérir progressivement le pouvoir un peu partout, en Europe et dans le monde.

Tout cela commande d’agir vite et fort. Or le moteur franco allemand est à la peine : la coalition outre Rhin vient d’imploser et nous savons combien notre pays, lui aussi, est fragilisé. Monsieur le ministre, quelle influence lui reste t il à

qu’il ne ferait finalement pas partie du nouveau collège. En moins de vingt quatre heures, l’Élysée a proposé la candidature de Stéphane Séjourné, ancien ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Le retrait tardif d’un candidat est inédit, s’agissant d’un grand pays comme le nôtre, et traduit une faiblesse certaine de la France, empêtrée depuis trois mois dans ses difficultés politiques internes et placée sous l’épée de Damoclès d’une procédure pour déficit excessif qui entame sa crédibilité. Dans le nouvel organigramme de la Commission, qui comprend, outre la présidente, vingt six commissaires, la place de la France a été préservée, en apparence, et même renforcée puisque Stéphane Séjourné serait nommé vice président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, alors que Thierry Breton n’occupait pas de poste de vice président. Toutefois, Thierry Breton disposait d’un très large portefeuille et exerçait, en pratique, une grande influence au sein de la Commission européenne. Le nouveau commissaire européen français, lui,

de plusieurs commissaires européens, mais ce rôle n’est pas très clair. Dans le nouvel organigramme, certains commissaires européens sont en effet placés sous la tutelle de plusieurs vice présidents, tandis que d’autres relèvent en même temps d’un vice président et directement de la présidente de la Commission européenne. En outre, la nouvelle composition du collège reflète les nouveaux équilibres en Europe, marqués par un basculement vers l’est. Ainsi, le commissaire européen polonais obtient le portefeuille stratégique du budget, à la veille du lancement des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel. La place des pays baltes est également remarquable. Le poste de haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a ainsi été attribué à la candidate estonienne et le nouveau poste de commissaire européen chargé de la défense et de l’espace au candidat lituanien. Le Sud n’est pas pour autant oublié. La candidate socialiste espagnole hérite d’un large portefeuille consacré à la transition verte, tandis que le candidat italien du parti de Giorgia Meloni sera chargé de la cohésion et des réformes, deux sujets majeurs. Le passage de trois à six vice présidents dans cette deuxième Commission von der Leyen risque en outre de diluer leur poids respectif et de les empêcher de contrebalancer le pouvoir de la présidente, qui s’en trouve augmenté. La Commission européenne reste pourtant, en théorie, un organe collégial, dont le président n’est que le. Mais le Mais le caractère pléthorique et très politique de la nouvelle Commission renforce le poids de sa présidente qui, privilégiant un mode de gouvernance très centralisé, se positionne en cheffe d’un « gouvernement de l’Europe » plutôt qu’en responsable d’une institution indépendante, chargée d’incarner l’intérêt général européen. Quelle sera la cohérence d’ensemble de son action ? Ainsi, le renforcement de la base industrielle et technologique de défense (BITD) sera t il confié au haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au commissaire européen chargé de la défense et de l’espace ou bien au commissaire européen chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle ? La réponse à cette question n’est pas dénuée d’importance, compte tenu des sensibilités différentes des États membres concernant l’industrie de défense et le lien transatlantique. Il en va de même concernant la question sensible de l’énergie nucléaire, sur laquelle les positions des commissaires divergent de manière préoccupante. On peut aussi s’interroger sur le portefeuille de certains commissaires, comme celui qui est à la fois chargé de l’énergie et du logement, alors même qu’on ne trouve aucune référence à ce deuxième domaine dans les traités européens de fait, il ne s’agit pas d’une compétence de l’Union. Tout cela appelle la plus grande vigilance de notre assemblée : il nous appartient de vérifier à la fois que les compétences des États membres, et donc les principes de subsidiarité et de proportionnalité, seront bien respectées et que l’action européenne européenne prendra mieux en compte les réalités de terrain et la diversité nationale. La commission des affaires européennes du Sénat examinera d’ici à la fin du mois des recommandations que deux de ses vice présidents et moi même lui soumettrons. En matière européenne, il faut absolument parvenir à faire mieux et moins. J’espère pouvoir compter sur votre soutien en ce sens, monsieur le ministre. Je m’apprête également à déposer une proposition de loi visant à instaurer un contrôle parlementaire sur la nomination des membres français dans plusieurs institutions européennes, à commencer par la Commission européenne.

d’outils de politique commerciale pour répondre aux mesures protectionnistes de la Chine ou des États Unis. C’est une Europe moins naïve qui est en train d’éclore, mais nous devons aller plus vite et plus loin.

nos partenaires européens. C’est ainsi que nous bâtirons notre influence pour mettre en œuvre cet agenda.

Au fond, la question qui nous est posée [est] : voulons nous lire l’histoire écrite par d’autres, [à savoir] les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois […] ? Ou est ce qu’on veut écrire l’histoire ?

L’Europe est mortelle. » Il appelait dans le même temps à bâtir une défense « crédible », une Union « plus souveraine et plus puissante ». Ces discours fondateurs ont été suivis d’actes. En témoigne le rôle clé joué par la France dans le plan de relance post covid, d’inspiration keynésienne, à l’échelle continentale, qui a été largement salué,

En témoigne encore la position centrale de la France dans la nouvelle définition de la taxonomie européenne incluant le nucléaire. Notre pays s’apprête d’ailleurs à battre son record d’exportation d’électricité. Là encore, nous avons pesé

Vous le savez aussi bien que nous, et vous avez d’ailleurs voté, comme notre groupe, pour Ursula von der Leyen, contrairement à eux. Dans ce combat que nous menons collectivement contre les extrêmes, il n’est plus possible d’avoir un visage à Bruxelles et un autre à Paris.

déjà évoqué les récentes victoires remportées ces derniers mois. D’autres dossiers, en cours et à venir, porteront la marque de notre influence. Notre position sur l’Ukraine n’a pas évolué depuis le début du conflit. Elle doit être celle de l’Union. Le Président l’a rappelé, nous avons un intérêt commun à ce que la Russie ne l’emporte pas. En parallèle, la victoire de Donald Trump doit conduire l’Europe à prendre son destin en main et à ne plus compter sur une aide importante des États Unis, notamment au sein de l’Otan et dans le cadre

Nous pesons contre l’Allemagne, qui plaide pour une signature rapide, sans modification ni compensation. La ministre de l’agriculture l’a rappelé il y a quelques jours : nous sommes frontalement opposés à cet accord. Sur le volet migratoire, c’est également la position française qui a été adoptée par le Conseil européen. En effet, sur demande, notamment, de la France, les ministres de la justice et de l’intérieur se sont accordés sur la nécessité de réviser la directive Retour de 2008. La France, l’Allemagne et l’Espagne ont également obtenu l’avancée de l’entrée en vigueur du pacte pour la migration et l’asile dès 2025. Sur la compétitivité, Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne (BCE), prône dans son rapport des réformes d’une ampleur inégalée et chiffre à 800 milliards d’euros par an le besoin d’investissements supplémentaires. Face au risque isolationniste et protectionniste des États Unis, l’Europe doit se défendre économiquement en investissant pour résister dans la guerre commerciale qui s’annonce.

Notre pays devra convaincre les États dits frugaux d’emprunter cette voie, comme nous l’avons fait pour le plan de relance post covid. En outre, face au risque de hausse des droits de douane lié à la nouvelle donne internationale, l’Allemagne pourrait se tourner davantage vers l’Europe afin de garantir la compétitivité de ses entreprises dans un contexte de croissance atone. Dans son rapport, Mario Draghi souligne enfin la nécessité, pour la survie des industries européennes de défense, de passer à des commandes communes et plaide pour des règles de préférence européenne.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par un hasard du calendrier, les changements institutionnels en cours au sein de l’Union européenne coïncident avec le retour au pouvoir de Donald Trump aux États Unis. Il est indéniable que cette situation modifie l’environnement politique et il est essentiel que nous prenions rapidement la mesure de cette nouvelle réalité afin d’adapter nos stratégies politiques. Le retour de Le retour de Donald Trump à la tête des États Unis pourrait avoir des répercussions significatives sur nos relations transatlantiques, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen Orient, mais aussi sur les mouvements conservateurs en Europe qui le soutiennent et l’imitent. Par ailleurs, les États Unis, sous la direction de M. Trump, pourraient modifier leur approche de sujets cruciaux tels que le commerce international, le climat et les relations diplomatiques. Face à ce renouvellement institutionnel, à la nomination des nouveaux commissaires européens et au retour de l’, l’agenda des politiques européennes doit non seulement être clair, mais également juste, inclusif, écologique et démocratique. l’Union européenne se montre unie si elle ne veut pas être effacée par les États Unis. Il est impératif que les pays membres parlent d’une seule voix, surtout dans un contexte où l’individualisme de certains États pourrait mettre à mal les fondements mêmes de notre union.

En ce sens, l’agenda stratégique élaboré par le Conseil européen a mis en exergue des points sur lesquels l’Union et la France doivent parachever leur travail et maintenir une dynamique d’amélioration. Nous devons travailler pour une Europe forte, sûre, prospère, libre et démocratique. Les pays européens doivent parler d’une seule voix, d’abord dans le domaine de l’environnement. Alors

Les catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes, et dont l’intensité et la violence sont exponentielles – je pense bien évidemment aux événements ayant eu lieu en Espagne au début du mois –, doivent constituer un moteur dans l’appréhension des risques de demain et nous inspirer des

Encore une fois, l’élection de Donald Trump laisse présager des conséquences géopolitiques fortes pour l’Europe. C’est pourquoi la coopération entre les membres de l’Otan doit se raffermir. Enfin, d’un point de vue économique, nous avons toujours à l’esprit l’Union gagne en compétitivité, en attractivité et en rayonnement en valorisant son marché et ses travailleurs. Des économies sociales de marché robustes seront le moteur de la réalisation de nos ambitions.

le domaine des politiques centrales de concurrence lui a échappé et son influence pourrait par conséquent s’en trouver limitée. De nombreux domaines de son portefeuille font en outre l’objet d’une « co supervision La France n’aura la main, semble t il, ni sur la défense et l’espace ni sur l’énergie. Elle devra constamment négocier avec ses homologues pour promouvoir son agenda industriel, sans capacité apparente à peser sur les négociations budgétaires à venir. Malgré cela, je reste convaincu que notre pays restera fort et mobilisé en faveur de cette union des peuples qui nous est si précieuse. La France saura faire valoir ses positions à l’échelon supranational et retrouver l’influence qui a toujours été la sienne. À l’échelle nationale, nous, sénateurs du groupe du RDSE, y veillerons.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Le Président de la République avait été clair lors des discussions avec Mme von der Leyen au moment de constituer la future Commission européenne : il voulait pour la France un poste de vice président de la Commission, lequel devait lui permettre de décliner ses priorités en matière d’autonomie stratégique et de souveraineté économique.

Un tel désaveu nous conduit naturellement à nous interroger sur le poids de la France au sein des instances européennes, en particulier de la Commission. Stéphane Séjourné a été auditionné cet après midi par les quatre commissions du Parlement européen compétentes,

couramment appelée BITD, car c’est un véritable enjeu de la future Commission européenne. L’industrie de défense française a le vent en poupe. L’Insee a constaté une nette amélioration du climat des affaires dans ce secteur depuis 2021, pour les raisons que l’on connaît. Face à la montée des tensions géopolitiques, l’Europe a a voulu bâtir une économie qui tend vers l’économie de guerre. Je rappelle que la BITD regroupe en France près de 2 000 entreprises. Les industries de défense ont bénéficié de l’émergence d’une demande spécifique, dans le cadre de l’aide matérielle fournie à l’Ukraine par la France et l’Union européenne. Selon le Kiel Institute, Paris a contribué à ce jour à hauteur de 2,69 milliards d’euros à l’effort de guerre en Ukraine. Vous le savez, notre BITD dépend de notre souveraineté, et réciproquement. Tout ce qui viendrait contraindre demain notre production et nos exportations dans le secteur serait susceptible de fragiliser durablement un secteur clé de notre économie et de notre sécurité.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que près de 100 millions d’Européens ont faim, qu’ils peinent à se chauffer et à se loger, Mme von der Leyen a décidé que, pour la première fois de son histoire, l’Union européenne n’aurait plus de commissaire à l’emploi et aux droits sociaux à sa place est nommé un commissaire « chargée des personnes, des compétences et de la préparation ». On passe là d’une logique collective de prise en charge politique de la question de l’emploi à une logique individuelle de responsabilité personnelle du rapport au travail.

La nomination d’Andrius Kubilius au commissariat à la défense a le mérite de lever les masques et relègue quelque peu le « mythe fondateur de la paix ». L’Union européenne semble se préparer à faire la guerre, tout en restant subordonnée à l’Otan. Sous la houlette des États Unis, nous avons intensifié notre production d’armement sur le continent, ainsi que le soutien financier et militaire à l’Ukraine. Pour quels résultats ?

chers collègues, la perte de maîtrise des conséquences de ce conflit se précise et, de ce fait, le spectre d’une troisième guerre mondiale se matérialise peu à peu. La dérive belliciste de l’Union européenne ne s’arrête pas à nos frontières à l’est de l’Europe. le Proche Orient, le Conseil européen, sous prétexte du « droit d’Israël à se défendre » et de « l’attachement de l’Union européenne à la sécurité d’Israël », décide de maintenir l’accord commercial de l’Union européenne avec Israël, ce qui équivaut de fait à une forme de cautionnement

par la Commission européenne, sur « l’interprétation erronée de la résolution 2758 des Nations unies par la République populaire de Chine » visait à mettre directement en cause le principe d’une seule Chine, et avec lui, l’ordre international d’après guerre. Plutôt que d’agir dans le sillage de la communauté internationale en choisissant les instruments de la diplomatie et de la coopération, le bloc des Vingt Sept continue sa dérive belliciste en multipliant ses visites navales et ses exercices d’entraînement militaire conjoints conjoints en mer de Chine méridionale. Les grands perdants de cette dérive, ce sont les peuples européens. La présidente de la Commission a en effet estimé que les États membres devraient investir dans les prochaines années plus de 500 milliards d’euros dans la défense. si la force des armes reste inévitable dans un monde écrasé par les dominations, le surarmement – car c’est de cela qu’il s’agit – n’a jamais conduit à autre chose qu’à l’abîme.

Selon nous, pour échapper au déclassement de l’Union européenne, nous devrions collectivement mettre en cause le concept de sécurité, lequel est uniquement fondé sur des dépenses d’armement, de défense ou d’infrastructures militaires. Nous devons cesser d’ignorer que les insécurités que les insécurités sanitaire, alimentaire, énergétique et climatique, ainsi que l’absence de partage réel de la gouvernance politique de la mondialisation, sont au cœur de tous les conflits et par conséquent à la racine de toutes les guerres. Notre pays devrait contribuer à ce réveil.

Monsieur le ministre, la nouvelle Commission qui se met en place portera une immense responsabilité celle de répondre, ou non, aux défis existentiels auxquels nous faisons face, au premier rang desquels figure l’urgence climatique. Force est de constater que la composition et les premières orientations de cette future Commission suscitent de profondes inquiétudes. La domination des forces libérales et conservatrices, notamment la nomination d’un commissaire d’extrême droite, est un des signaux préoccupants. Le morcellement du portefeuille environnemental et la subordination apparente du Pacte vert pour l’Europe aux impératifs de compétitivité industrielle font craindre un recul de l’ambition climatique européenne, alors

que de l’autre côté de l’Atlantique, le président américain doute du changement climatique et a déjà annoncé vouloir, de nouveau, sortir de l’accord de Paris, l’Europe et la France

Dans ce contexte, la question de l’influence française prend une dimension particulière. La France ne peut se contenter de célébrer l’obtention d’une vice présidence exécutive, au portefeuille flou, sur la stratégie industrielle. Cette approche fondée sur le placement de candidats, fait du prince, et la défense de nos seuls intérêts industriels est dépassée ! Notre influence doit se réinventer. La France doit être la force motrice d’une réorientation écologique et sociale de la Commission. Concrètement, cela signifie qu’il faut porter trois exigences fondamentales. Premièrement, la Commission doit être la garante de l’ambition environnementale européenne et non pas son fossoyeur. Nous ne pouvons accepter que le Pacte vert soit vidé de sa substance au nom de la compétitivité. La France doit défendre l’exigence d’objectifs climatiques contraignants, d’une sortie effective des énergies fossiles et d’une protection réelle de la biodiversité. la transition écologique doit être socialement juste. Exigeons un fonds social climat réellement doté et des mécanismes efficaces de solidarité européenne ! Troisièmement, la France doit défendre une vision de l’Europe comme projet politique, démocratique et fédéral, et pas seulement comme marché ou puissance industrielle. La question du Mercosur illustre parfaitement ces contradictions. Vous avez sans doute lu, monsieur le ministre, la tribune adressée aujourd’hui par plus de six cents parlementaires français à Ursula von der Leyen, dans laquelle ils indiquent que les conditions d’un accord ne sont aujourd’hui pas réunies.

Cette tentative de passage en force portant sur un accord aux conséquences environnementales désastreuses est grave ! Elle créerait un précédent dangereux en matière de gouvernance européenne, tout en encourageant la déforestation en Amazonie et le développement d’une agriculture intensive incompatible avec nos objectifs climatiques. Si la Commission s’engageait dans cette voie, elle n’affaiblirait pas seulement la position française : elle saborderait sa propre crédibilité en matière de lutte contre le changement climatique et de respect des opinions publiques du continent. d’autonomie stratégique européenne, le soutien à l’Ukraine est une nécessité absolue. Nous devons maintenir notre engagement à ses côtés face à l’agression russe, particulièrement dans la période d’incertitude qui s’ouvre concernant le soutien des États Unis. Nous avons aussi besoin d’une vision plus large de la sécurité européenne, qui intègre pleinement les enjeux climatiques, alimentaires et sanitaires. La première des autonomies est énergétique c’est en accélérant le développement des énergies renouvelables que nous renforcerons véritablement notre indépendance. Une Europe qui continuerait à subventionner les énergies fossiles ferait fausse route. Face à un président américain climatosceptique, qui menace d’imposer des droits de douane punitifs et de saper l’alliance transatlantique, l’Europe doit plus que jamais affirmer son autonomie, sa solidarité et ses valeurs, dans le cadre d’un véritable projet politique alternatif : celui d’une Europe qui protège ses citoyens et son environnement, qui investit massivement dans la transition écologique, qui renforce sa cohésion sociale face aux menaces externes. Les tensions commerciales annoncées avec les États Unis doivent être l’occasion d’accélérer notre transition vers une économie décarbonée et circulaire, et non pas de renoncer à nos ambitions environnementales. L’Europe ne peut plus se permettre d’être suiviste. C’est à cette condition que l’influence française retrouvera son sens, non pas comme une fin en soi, mais comme un levier au service d’une transformation profonde de l’Europe. La France a une responsabilité historique, celle de montrer qu’une autre Europe est possible : une Europe de la transition écologique, de la justice sociale, du respect des droits fondamentaux, de la justice internationale et de la démocratie vivante. C’est ce message que je vous invite à porter avec force lors de vos discussions avec la nouvelle Commission sur les chantiers à venir à l’échelon européen.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment de l’installation de cette nouvelle Commission, nous sommes, pour notre part, prêts à travailler dans un esprit de compromis, celui qui caractérise nos institutions européennes. Cependant, nous sommes inquiets.

Cette alliance s’accompagne d’un virage sécuritaire et d’une présidentialisation de la cheffe de la Commission, qui a divisé les portefeuilles de ses commissaires et écarté tout profil susceptible de faire contrepoids à son autorité. Les partis conservateurs, apparemment fermement pro européens, mettront ils en cause le projet qui doit nous unir ? Le risque est celui d’un détricotage des législations européennes les plus ambitieuses – nous pensons notamment au récent Pacte vert au récent Pacte vert – et des dernières avancées. Alors qu’à la suite de l’épidémie de covid 19, l’Europe de la santé émerge à peine, la présidente de la Commission abandonne ces questions à un proche de Viktor Orban, qui ne dispose d’aucune expérience sur le sujet. Pis, la présidente souhaite intégrer le programme EU4Health au sein d’un grand fonds de compétitivité, actant la prévalence des logiques de rentabilité sur celles de santé. Cette impulsion vers un capitalisme financiarisé nous inquiète. En matière de migration, la dynamique tend clairement vers un durcissement des politiques européennes. La Commission souhaite passer de nouveaux accords avec des pays tiers pour la gestion des centres d’asile. Or de tels centres existent déjà en Tunisie, en Libye, en Turquie de nombreuses violations des droits humains y ont été constatées. La présidente de la Commission et son commissaire aux affaires intérieures et à la migration appuient l’accord contesté entre l’Italie et l’Albanie, malgré son invalidation par les tribunaux italiens et l’avis des tribunaux européens. En choisissant de généraliser l’externalisation de la gestion des migrations, l’Union européenne se défausse de ses responsabilités. Elle ferme les yeux sur les violations des droits fondamentaux qui sont commises en dehors de son territoire. Pourtant, la Commission avait elle même pointé en 2018 les risques légaux liés à l’utilisation des centres de retour. Elle notait un risque élevé d’enfreindre le principe de non refoulement et soulevait des doutes quant à la conformité de ces centres aux valeurs de l’Union. Or, aujourd’hui, ces valeurs mêmes sont remises en cause. Pour notre part, nous souhaitons préserver l’acquis européen et défendre un modèle autre que celui du repli sur soi et du rejet de l’autre. Mais, pour ce faire, encore faut il avoir une voix. voix. Force est de constater que la France n’arrive plus à faire entendre la sienne au sein de l’Union européenne. Notre perte d’influence, illustrée par la mise à l’écart autoritaire de Thierry Breton, a déjà un effet visible à l’échelon européen.

France est aujourd’hui plus isolée que jamais. Le couple franco allemand, locomotive historique de l’intégration européenne, est désormais doublé par une Europe dont le pivot glisse inexorablement vers l’est. Par ailleurs, il nous faut bien constater que ces dernières années la France a trop souvent soutenu des positions relativement souverainistes, contre la logique de compromis. Elle est apparue comme défendant trop fréquemment ses seuls intérêts propres. Ce faisant, elle a perdu de sa capacité à fédérer, à créer ce consensus qui est si fondamental dans le projet européen.

Enfin, les résultats des élections outre Atlantique nous rappellent notre besoin vital d’une Europe forte et indépendante. Nous sommes désormais un peu plus seuls en tant qu’Européens, car le président Trump n’est pas, et ne sera pas, un ami de l’Europe. Le retour de la guerre, la compétition internationale, la relocalisation des industries, l’effondrement climatique sont autant de défis qui ne peuvent appeler qu’une réponse commune. Aucun de ces sujets ne sera résolu par les égoïsmes des nations. Aussi, il est d’autant plus important de développer des politiques fortes, de réaffirmer nos valeurs, notre attachement à l’Europe sociale et à la démocratie. L’Europe est capable de s’ériger en modèle de référence. Il faut qu’elle le veuille ; pour notre part,

l’on aime ou que l’on déteste Donald Trump, une chose est tout à fait certaine : il aura pour seule boussole la défense des intérêts américains. Trump ne nous fera pas de cadeaux. Alors, le meilleur cadeau que nous pouvons nous faire, à nous Européens, c’est de ne pas lui en faire Il s’agit non pas d’ouvrir les hostilités avec nos alliés historiques, mais d’adapter notre positionnement stratégique à cette nouvelle donne géopolitique. L’Union européenne doit redevenir une puissance si elle ne veut pas rester la vassale des autres puissances. Elle doit rester fidèle à ses valeurs et s’engager pour la paix et la prospérité, mais elle doit surtout défendre ses intérêts. Le déclin géopolitique du vieux continent s’explique d’abord par son décrochage économique. Pour redevenir une puissance, l’Europe doit renouer avec la croissance. Pour ce faire, elle doit redevenir une terre de production. J’identifie trois principaux chantiers pour y parvenir : investir massivement dans l’innovation ; mobiliser la commande publique pour nos entreprises ; faire de l’action climatique un levier de compétitivité. Premier chantier : pour rester dans la compétition technologique mondiale, l’Europe doit faire de l’innovation une obsession économique. C’est non pas une option tactique pour tenter de gagner une ou deux places dans la compétition mondiale, mais une question de vie ou de mort. Si nous cessons d’innover, nous ne pourrons plus garantir la pérennité de notre modèle socio économique. Il fallait sans doute qu’un Européen convaincu le dise aussi crûment pour que tous les Européens commencent à y croire. En effet, le rapport Draghi est très clair : si nous n’investissons pas massivement pour moderniser notre économie, l’Union européenne ne pourra plus justifier sa propre existence. Mario Draghi estime cet effort à 800 milliards d’euros par an. Comment administrer un tel électrochoc ? À l’évidence, il faut précisément moins administrer. La bureaucratie ne favorise jamais la compétitivité j’y reviendrai. La puissance publique dispose aussi d’un puissant levier d’action pour servir en priorité les intérêts européens : la commande publique. La révision de la directive de 2014 sur la passation des marchés publics doit permettre une réorientation stratégique claire. Nous devons donner priorité à nos entreprises. Pour appréhender la mondialisation avec un peu plus de sérénité, il faut cesser de considérer que les Européens sont des consommateurs avant d’être des producteurs. troisième chantier consiste à faire de l’action climatique un levier de compétitivité, et non l’inverse. Le Pacte vert de la précédente Commission partait d’une excellente intuition : la pérennité de notre économie passe par la transition écologique, simple raison que le réchauffement climatique menace nos intérêts économiques. Mais la transition écologique ne doit être ni un exercice de repentance ni un appel à la décroissance. Le Pacte vert, par sa dérive bureaucratique, risque de plomber notre économie. ce propos par un sujet cher à mon cœur : l’agriculture. Celle ci ne saurait être la seule priorité de la nouvelle Commission, mais elle sera la jauge de son succès. Si l’Europe continue à ouvrir ses marchés à tous les vents, tout en étouffant ses propres agriculteurs sous les normes, alors elle aura échoué.

En outre, le rapport Draghi identifie de nombreuses pistes prioritaires comme l’unification des marchés de capitaux, l’union bancaire, la réforme de la politique de concurrence et des aides d’État, la simplification et le soutien à l’innovation

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous débattons ce soir de la politique européenne de la nouvelle Commission et de l’influence de la France, il me semble important d’aborder notre politique étrangère et certains de ses corollaires en ayant en tête l’agitation internationale. La nouvelle Commission européenne doit inspirer à la France de la vigilance, de l’exigence et de l’anticipation. Tel n’a malheureusement pas toujours été le cas dans le passé… Tout en restant fidèle à ses engagements européens, la France a des intérêts à défendre. La nouvelle Commission, elle, doit entendre les États membres et ne pas donner l’impression de naviguer à vue.

Poser la question, c’est commencer à y répondre. Anticipons avec lucidité. Oui, la France doit faire entendre sa voix et tempérer un tropisme qui, en l’état, ne sert pas suffisamment ses intérêts.

En tant qu’Européens, nous ne pouvons ignorer la fragilité de notre autonomie stratégique et notre besoin de maintenir une alliance transatlantique équilibrée. Au milieu des turbulences mondiales, nous ne devons pas oublier nos rivaux géopolitiques que sont la Chine, la Russie ou encore l’Iran. Les États Unis seront toujours fidèles à eux mêmes et nos attentes ne sauraient être démesurées. Soyons réalistes et pragmatiques, car aucune des deux dernières administrations américaines n’était plus favorable que l’autre à l’Europe.

Plus généralement, ces règles sont allées dans le sens d’une limitation du monopole des grandes plateformes, en imposant des règles de transparence à leurs algorithmes.

harmonisées concernant l’intelligence artificielle adopté cette année a permis de définir un cadre rigoureux pour garantir que les IA soient sûres, transparentes et respectueuses des droits fondamentaux. Des restrictions ont été prévues pour les systèmes à haut risque, comme ceux qui sont utilisés dans les domaines de la reconnaissance faciale ou du recrutement. Malheureusement, ce règlement ne fait qu’effleurer le sujet et de lourdes incertitudes demeurent, notamment dans le volet relatif l’IA est de plus en plus implantée dans ce domaine, la nouvelle Commission devra remettre l’ouvrage sur le métier. Il est urgent de permettre l’émergence de solutions cybereuropéennes et indépendantes. De même,

Il y a urgence à agir, car les géants du numérique outre Atlantique battent tous les records d’investissement dans l’intelligence artificielle, sur fond d’une compétitivité déjà asymétrique entre l’Europe et les États Unis. En conclusion, En conclusion, qu’il s’agisse de grande diplomatie ou de, la nouvelle Commission ne peut se permettre d’osciller entre navigation à vue et absence de vision à long terme. Plus que jamais, la vigilance, l’exigence et l’anticipation doivent être de mise. Monsieur le ministre,

Pour accroître l’innovation, il est proposé de doubler le budget du programme cadre de recherche et d’innovation en le portant à 200 milliards d’euros sur sept ans et de créer une agence européenne pour l’innovation. Cette mesure va dans le bon sens. Nous avons en Europe des ingénieurs et des chercheurs de talent ; encourageons les à rester chez nous et à ne pas céder aux sirènes des géants américains du secteur. Garder les talents européens sur le sol européen,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la nouvelle Commission, plus conservatrice que jamais, devra pourtant reprendre le chantier le plus ambitieux de notre histoire, celui du Pacte vert.

où la nature périclite, où les sols s’appauvrissent, où le climat s’emballe et où les catastrophes s’enchaînent. Pourtant, alors que les circonstances exigent de faire preuve de volontarisme, la composition politique de la nouvelle Commission ne reflète en rien les préférences électorales des citoyens. Tout concourt à faire d’elle un simple secrétariat du Conseil européen, dénué de toute autonomie et incapable de définir un intérêt général. La Commission étant dominée par des gouvernements réactionnaires, la culture européenne du consensus est dangereusement mise en péril. La Commission ne doit pas céder à la pression politique des extrêmes. L’Union européenne doit rester ce lieu où nous faisons en conscience des choix inscrits dans le long terme pour le climat, pour une alimentation durable, pour la biodiversité et pour plus de justice.

Or rien n’est plus délétère que l’incertitude provoquée par les atermoiements et les renoncements qui brouillent notre message et nous détournent de ce que nous sommes. Le fameux cap devient un chemin en zigzag, l’objectif s’éloigne et le découragement, voire le cynisme, nous gagne.

La révision du règlement Reach, pierre angulaire de la stratégie « zéro pollution », a également été reportée à plusieurs reprises. Enfin, les ambitions environnementales de la politique agricole commune (PAC), fruits de plusieurs années de travail et de réflexion, ont été enterrées en l’espace de quelques semaines, que le projet d’interdire la vente de moteurs thermiques d’ici à 2035 suscite déjà une fronde. Le retour de Donald Trump sur la scène internationale signifie en outre le mépris des règles, la défense coûte que coûte des énergies fossiles, l’entrave à la

Aux plus conservateurs d’entre nous, à ceux qui demeurent attachés à la préservation de la nature et des paysages, qui renvoie à une tradition, à une identité, à un modèle d’agriculture familiale, à une alimentation locale, je demande de ne pas oublier cette fameuse phrase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa Si nous voulons que rien ne change, il faut tout changer. » Que nous le voulions ou non, le monde est en mutation. Notre responsabilité, celle de la France dans une Union incertaine et imprévisible,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, et si nous passions à l’âge adulte ?

presque aveuglément leur sécurité au parapluie américain. Par conséquent, nous avons un rôle particulier à jouer pour aller vers l’autonomie stratégique.

placent la relation transatlantique au cœur de leur sécurité. Sachons répondre à leurs inquiétudes et à leurs préoccupations géopolitiques : c’est ainsi que nous pourrons bâtir l’Europe de la défense, l’autonomie stratégique et la souveraineté européenne que nous appelons de nos vœux.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par un curieux hasard, l’installation de la nouvelle Commission européenne intervient au même moment que l’élection d’un nouveau président aux États Unis.

président de la commission des affaires européennes du Sénat, notre collègue Jean François Rapin, a parlé à juste titre de réciprocité et de préférence communautaire, ces principes semblant toujours oubliés dans les discours européens.

ne nous défaussons pas en pensant que les seules difficultés viennent de l’extérieur. Elles sont aussi le fruit de problèmes endogènes, d’un manque de vision et d’une absence d’ambition.

au risque, sinon, de créer une fracture définitive et irrémédiable. Chaque pays européen pourrait alors être tenté de faire bande à part. Nous n’avons pas besoin de cela. Une Europe qui protège est aussi une Europe qui entreprend et qui avance, dans un monde qui sera celui de la revanche du Sud global.

par celui de la compétitivité, de la productivité et de la prospérité de notre continent, qui sera au cœur du portefeuille de notre commissaire Stéphane Séjourné. Nous devons nous donner les moyens de mobiliser l’épargne publique et privée pour investir massivement dans l’innovation, dans la technologie,

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, il me revient la tâche de conclure ce débat – lourde tâche que de conclure après la conclusion

en raison d’un contexte politique interne très différent de celui de 2019, qui se reflète à la fois dans la composition du nouveau Parlement européen et dans celle du Conseil européen. Dans les deux cas, on observe un net déplacement du centre de gravité des institutions européennes vers la droite et, pour ce qui concerne le Parlement, une montée inquiétante des mouvements nationalistes. Elle s’en distingue ensuite en raison d’un environnement international également très différent de celui de 2019, instable et globalement hostile, marqué par la guerre en Ukraine, les événements du Proche Orient, la menace économique et géostratégique chinoise et la prochaine installation d’une administration américaine protectionniste. Il en découle une réorientation des priorités de la Commission. S’il est toujours question de poursuivre un agenda environnemental et numérique ambitieux et de conserver un certain attachement de l’Union européenne au multilatéralisme, dans la sphère internationale, ces thèmes cèdent à présent le pas à des objectifs de compétitivité, de croissance, d’emploi, de réindustrialisation, d’autonomie stratégique, économique et militaire et, plus généralement, de défense résolue des intérêts européens dans tous les domaines. nombre de mes collègues viennent de le souligner. Pour ma part, je me réjouis de ce nouveau souci de réalisme affiché par la Commission. Reste à voir si la cohésion des États membres et les moyens mis en œuvre seront suffisants pour que de réels progrès puissent être enregistrés sur tous ces sujets,

Elle inquiète ses partenaires par les déficits qui plombent ses finances publiques : « une nation qui ne tient pas ses comptes ne peut pas tenir Par ailleurs, comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner dans cet hémicycle, notre pays me paraît aujourd’hui très affaibli dans chacune des grandes institutions européennes. Au Conseil européen, il est représenté par un Président de la République qui non seulement ne pourra se représenter en 2027, qui a de surcroît subi, à travers les partis qui se réclament de lui, deux échecs électoraux successifs, lesquels lui ont fait perdre une bonne part de sa crédibilité aux yeux de ses homologues européens. Au Conseil des ministres de l’Union européenne, notre pays est représenté par un gouvernement de compromis, que je soutiens, mais dont l’assise parlementaire est fragile et qui doit assumer à Bruxelles comme à Paris une situation budgétaire très dégradée, comme je viens de le dire, privant la France de réelles marges de manœuvre politiques.

insuffisamment qualifiée à mon sens pour exercer des responsabilités de ce niveau. Le putatif commissaire français se trouve certes paré d’un beau titre de vice président exécutif,

et sur la capacité de la France à peser sur les décisions importantes qui devront être prises. J’espère, bien évidemment, en tant que Français et Européen convaincu, que les faits me donneront tort.